La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 11 mars 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la sécurité globale

Merci, Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me présenter devant la Haute Assemblée pour évoquer cette proposition de loi

ces polices municipales et les maires concourent à la sécurité de nos concitoyens, ne serait-ce que pour appliquer les arrêtés du maire, qu'ils soient relatifs à la tranquillité ou à la salubrité publiques.

Il ne s'agit pas de faire à la place de l'État, mais il ne s'agit pas non plus de donner des pouvoirs de police judiciaire aux polices municipales. En effet, si nous donnions des pouvoirs de police judiciaire aux polices municipales,

(CNIL) a considéré que le législateur n'avait pas épuisé sa compétence et qu'il aurait dû légiférer sur l'utilisation des drones.

d'autres façons de faire pour mutualiser les moyens d'intervention. Une disposition permet ainsi, sur le modèle de ce qu'a proposé le conseil départemental de l'Oise, de relier des caméras de vidéoprotection à un centre de supervision urbain en lien direct avec le département et non plus avec la commune ou l'agglomération.

Après les polices municipales et les images, le troisième sujet est la sécurité privée. La sécurité privée est partout sur le territoire national.

très utile : plus personne aujourd'hui n'imagine qu'un grand magasin soit tenu par des policiers, chacun comprenant que c'est un agent de sécurité privée qui organise cette sécurité.

à la sécurité de nos concitoyens. Le quatrième sujet est la protection que nous devons aux forces de l'ordre, aux femmes et aux hommes qui, tous les jours, risquent leur vie pour nous protéger dans des conditions que nous savons de plus en plus violentes et difficiles, parce que la société est de plus en plus violente

toute la volonté du ministère de l'intérieur et du Gouvernement de maintenir une disposition qui n'a rien à voir avec l'article 18 de la loi dite « Séparatisme », en ce sens qu'il vise à protéger les policiers et les gendarmes au cours des opérations de police.

Il ne s'agit pas pour le Gouvernement, en soutenant la proposition de loi de l'Assemblée nationale, d'imaginer une police fédérale et une police locale. Ce n'est pas souhaitable un seul instant, mais nous ne souhaitons pas non plus

Vous l'avez dit, monsieur le ministre, la proposition de loi relative à la sécurité globale a connu diverses péripéties qui ont induit beaucoup de confusion et d'inquiétude, alors même qu'elle comporte de nombreuses dispositions intéressantes visant à faciliter la complémentarité de l'action des différentes composantes de la sécurité intérieure de notre pays. Je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot

Mais nous avons tous noté que cette proposition a été retirée, que le ministère de l'intérieur s'en est saisi et que le texte comporte désormais des propositions beaucoup plus importantes et structurelles, que vous avez commentées à l'instant.

la saisine préalable du Conseil d'État et la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Pourtant, ces études et saisines auraient pu éviter bien des polémiques.

Prenant acte de la montée en puissance des polices municipales, l'article 1 de la proposition de loi prévoit d'élargir, à titre expérimental, les prérogatives judiciaires des agents de police municipale sous l'autorité du parquet fonctionnel et toujours sous l'autorité hiérarchique du maire. En 2011, le Conseil constitutionnel a posé deux limites à l'extension de ces prérogatives, en indiquant qu'elles devaient être exercées sous l'autorité du procureur et que les policiers municipaux ne pouvaient bénéficier de pouvoirs généraux ni d'enquête ni d'investigation. Nous nous sommes donc tenus à cette ligne rouge.

donc davantage du bon sens que d'une volonté de changer la durée de l'expérimentation, que vous aviez prévue plus courte, je suppose, dans un souci d'aller plus vite.

les cigarettes de contrebande, mais aussi les défauts de permis de conduire et, donc, la saisie de véhicules. Or nous n'avons pas à ce jour de réponse satisfaisante des administrations centrales quant aux conditions de cette saisie.

Vous nous avez proposé une nouvelle rédaction visant à réprimer la provocation à l'identification des policiers, gendarmes et policiers municipaux. Enfin, l'article 23 revoit complètement le régime des réductions de peines. Au total, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons essayé de dépassionner ce débat

loi renforce la complémentarité entre les différents acteurs de la sécurité, grâce à des dispositions sur la sécurité privée et sur la sécurité dans les transports, auxquelles je me suis plus particulièrement intéressé. J'évoquerai également le volet relatif à la vidéoprotection et à la captation d'images, destiné à amplifier les moyens d'action dont disposent nos forces de sécurité. Sur ces différents points, la commission des lois s'est attachée à conserver les apports

Le texte entend mieux encadrer le recours à la sous-traitance dans les activités de surveillance et de gardiennage. Il renforce également les prérogatives du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps), qui assure la police administrative du secteur. Ses agents de contrôle pourront notamment constater par procès-verbal certaines infractions. La proposition de loi vise aussi à garantir la qualité du recrutement et de la formation des agents privés de sécurité. Si la commission partage cet objectif, elle a veillé cependant à ne pas exclure du marché du travail des personnes peu qualifiées qui trouvent dans les métiers de la sécurité une première opportunité d'embauche et, donc, une première expérience professionnelle. En contrepartie de cet effort de professionnalisation, le texte prévoit de confier de nouvelles responsabilités aux agents privés de sécurité, mais de manière très ponctuelle, comme nous aurons l'occasion de le voir au cours du débat.

pas refuser le progrès technique quand il sert l'efficacité des forces de l'ordre, il convient de toujours vérifier que ces innovations ne menacent pas les libertés publiques, auxquelles nos concitoyens comme nous-mêmes sommes légitimement attachés. La commission a tenu à s'assurer que les captations d'images répondent à des nécessités opérationnelles précises, que les finalités soient bien établies, que la formation des personnels destinataires de ces images soit suffisante, que la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès soient bien garanties.

concerne les caméras mobiles des forces de l'ordre, nous avons refusé la diffusion d'images directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux, car elle risquerait d'alimenter ce que nous avons appelé- c'est vrai, monsieur le ministre -la « bataille médiatique » ou la « guerre des images au lieu d'apaiser les relations entre la police et la population, ce qui doit être notre première préoccupation. Nous avons également limité à des motifs opérationnels précis la possibilité de consultation immédiate par les agents des images de leurs caméras mobiles.

avons menés avec Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. En conclusion, mes chers collègues,

interviennent dans ce domaine, dont : les douanes, la brigade des réseaux franciliens, la police aux frontières, le groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) pour la RATP, la SUGE pour la SNCF, des entreprises privées, et parfois d'autres.

national du maintien de l'ordre ; d'autre part, le Livre blanc de la sécurité intérieure, qui préfigure une troisième loi pour la programmation de la sécurité intérieure, après celles de 2002 et de 2009. Pourtant, loin de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens en matière de sécurité, les politiques gouvernementales menées depuis 2002 en faveur du « tout-sécuritaire » se sont toutes révélées contre-productives. Ce projet de société mûri depuis de nombreuses années arrive à un point de maturation important. En effet, le

la délégation des missions de services publics à des entreprises qui n'ont pour unique finalité que la recherche de la rente. En parallèle, on se dote d'outils de surveillance massive, toujours plus prégnants sur notre territoire.

Tous les dispositifs qui y figurent ont en commun d'augmenter la surveillance et la répression dans l'espace public. Plusieurs libertés sont ainsi mises en péril, telles que celle d'aller et venir anonymement dans l'espace public,

qui conduira les populations à « s'autocensurer ». En outre, cet usage disproportionné de nouvelles technologies porte atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles comme l'a, à plusieurs reprises, rappelé la Cour

la rédaction reste si floue qu'elle laisse toujours une latitude importante pour réprimer tout comportement visant à dénoncer des actes commis par les forces de l'ordre et, donc, pour limiter ainsi la possibilité de contestation au profit d'un pouvoir de police fort et indiscutable.

invisibilise » toute dérive. Il ne s'agit en aucun cas de protéger les policiers, mais d'empêcher toute diffusion d'image compromettante. Mes chers collègues, ce texte acte un changement de paradigme en matière de sécurité publique. L'espace public devient un espace de contrôle et de suspicion où chaque citoyen est considéré comme un suspect, voire un terroriste potentiel, en tout cas comme une menace.

Nous sommes bien loin de la tradition française du maintien de l'ordre par la désescalade de la violence. On assiste au contraire à un déferlement de violence, ces dernières années, contre le mouvement social en particulier. En défendant ce texte, le Gouvernement fait la démonstration de son incapacité à penser la police dans notre démocratie. Depuis des décennies, on met bout à bout « plusieurs polices » sans réévaluer le système dans son ensemble. La question des valeurs n'est pas

Un vrai texte de sécurité globale ne devrait-il pas contenir des mesures sur le logement, l'éducation, l'alimentation, la santé ?

on recule sur les libertés. Nous considérons que la lutte contre l'insécurité exige la mobilisation de l'ensemble des services publics et leur développement dans tous les territoires de la République. Le récent rapport sur la pauvreté en France, publié par l'Observatoire des inégalités, est une illustration dramatique des inégalités territoriales. C'est sur ce terreau de la disparition des services publics que se développent les trafics de stupéfiants et la loi des bandes organisées.

Représente-t-elle une possibilité d'évolution positive ? Bien sûr que oui ! Mes chers collègues, c'est notre devoir de voter contre cette motion de rejet que propose la gauche de la gauche de notre hémicycle. Cette gauche qui estime que les voyous ont toujours des excuses atténuantes et les forces de sécurité toujours des circonstances aggravantes.

qui, le 12 novembre 2018, s'est donné la mort, anéantie par le harcèlement et les menaces qu'elle subissait. Oui, nous, sénateurs Républicains, avons pleuré Mélanie Lemée, cette jeune gendarme de 26 ans, fauchée volontairement le 4 juillet 2020 par un chauffard. Nous aussi ! Oui, nous, sénateurs Républicains, avons une pensée en ce moment pour ce jeune policier et sa compagne policière, assassinés chez eux, à Magnanville, le 13 juin 2016 devant leur jeune fils de 3 ans. La tergiversation n'est pas de mise face au sacrifice du colonel Arnaud Beltrame, que nous ne devrons jamais oublier. Insultes, crachats, coups et blessures, menaces de mort, tel est le triste quotidien que vivent de nombreux gendarmes et policiers, dans le silence médiatique le plus absolu. L'état moral de ces femmes et de ces hommes, qui servent la République au quotidien, ne cesse de s'aggraver. Notre devoir est de leur donner les moyens de lutter concrètement contre cette violence qui ne cesse de s'intensifier. Alors qu'ils risquent leur vie pour assurer notre sécurité, la réponse pénale face aux délinquants se révèle très souvent, trop souvent, insuffisante, pour ne pas dire dérisoire. Ce constat est terrible, car il traduit le sentiment d'abandon et de mépris que subissent nos policiers et nos gendarmes, qu'ils ressentent au tréfonds d'eux-mêmes. Mes chers collègues, je vous le dis, tout ce qui peut être voté pour assurer la sécurité des Français et la protection de ceux qui en sont les garants est une excellente chose. S'y opposer, c'est mettre encore plus en péril leur sécurité et même leur intégrité, leur honneur, leur famille, bref, leur environnement de vie professionnel et privé. Alors que les crimes violents se multiplient et que nos forces de sécurité se retrouvent de plus en plus souvent dans des situations extrêmement difficiles dans l'exercice de leur métier, nous devons absolument être à leurs côtés Pour conclure, je voudrais inviter ceux qui ont cosigné cette motion à faire une visite de l'établissement de santé Le Courbat, qui accueille les agents en dépression, en burn-out ou tout simplement épuisés, détruits physiquement et psychologiquement. Oui, nous y avons été et nous avons constaté Allez-y, vous comprendrez la détresse de leur famille, l'angoisse que ces femmes et ces hommes vivent au quotidien ! Quel c'est sans hésiter une demi-seconde que je vous demande de voter contre cette motion de rejet, pour dire aux forces de sécurité que nous les respectons, que nous les soutenons dans leur travail et que nous légiférons pour les aider à faire face. La Haute Assemblée sortira grandie et se montrera pleinement responsable si elle sait prendre la juste mesure de cet important dossier que constitue la sécurité publique. Sans sécurité, il n'y a plus de liberté. Les Françaises et les Français espèrent nous voir enfin donner des moyens et des compétences élargies aux forces de sécurité intérieure pour assurer la quiétude publique, qui disparaît un peu plus chaque jour.

En effet, on pouvait espérer qu'une proposition de loi, encore intitulée « sécurité globale », s'attelle d'abord à améliorer les conditions de travail et la formation des policiers, à lutter contre le mal-être de nombreux agents, à renforcer les équipes, dans la sérénité une confiance entamée entre la France et sa police, à exiger une police exemplaire qui protège en luttant avec fermeté contre toutes les dérives, même marginales, qu'il s'agisse de violence, d'actes de racisme ou de sexisme, à créer une autorité indépendante de contrôle de la police pour lutter contre l'impunité, l'impunité, à revoir une doctrine de maintien de l'ordre qui, trop souvent, tue et mutile des manifestants, à réinvestir les quartiers populaires en créant une véritable police de proximité. Rien de tout cela ! À la place, on nous propose un désengagement massif de l'État, qui se défausse de ses responsabilités sur les polices municipales et la sécurité privée, désengagement qui porte en germe un renforcement dramatique des inégalités territoriales, une course à l'armement qui s'apparente à une véritable fuite en avant sécuritaire, une dérive orwellienne de surveillance de masse, qui, avec le funeste article 24 notamment, piétine les droits des individus et les libertés publiques, au premier rang desquels la liberté d'informer et le droit de manifester. On ne peine guère à trouver outre-Atlantique le modèle qui vous inspire, et il fait froid dans le dos ! Une image glaçante vient à l'esprit : celle de ces polices municipales américaines, plus équipées que des soldats, moins formées que des réservistes de la gendarmerie, qui abattent dans le dos des citoyens en fuite, le plus souvent afro-américains. Naturellement, cette perspective effrayante nous est proposée par un ancien chef du RAID, sans avis du Conseil d'État ni étude d'impact, le tout en plein état d'urgence sanitaire, alors que le droit de manifester est contraint, et ce contre l'avis de toutes les associations de défense des libertés publiques ou de la Défenseure des droits. N'en jetez plus, la coupe est pleine ! Alors que la crise sanitaire dure et nous épuise, que la crise économique et sociale s'aggrave jour après jour, qu'il nous faut inventer le monde d'après, sobre et résilient, le Gouvernement n'a rien d'autre à proposer aux Françaises et aux Français que la poursuite de cette dérive sécuritaire et liberticide.

La police de la République est issue de la République. D'ailleurs, cher Henri Leroy, sur ces travées, nous sommes tout aussi attachés à la sécurité des policiers et des gendarmes que vous.

C'est précisément la raison pour laquelle nous allons développer des arguments dans ce débat. Il nous semble que, en guise de continuum, vous nous proposez une confusion. Tout le monde va tout faire, mais personne ne va rien faire correctement, et pas partout ! Les polices municipales sont inégalitaires, parce que toutes les municipalités n'ont pas les mêmes moyens.

aurait mérité, à mon sens, d'être examinée en même temps que le prochain projet de loi confortant le respect des principes de la République, car il existe une osmose entre ces deux textes.

qui jouent un rôle très semblable à celui des policiers municipaux. C'est un exemple parmi d'autres : de nombreux autres services de l'État ou services parapublics

la police a finalement moins de pouvoirs que les douanes. Dans d'autres cas, c'est bien entendu l'inverse. Plus généralement, il faut bien voir que, face à la délinquance,

plus de la moitié de nos concitoyens se sentent en insécurité au quotidien. Cette triste réalité est reflétée par un sondage paru en fin d'année dernière, mais aussi par l'actualité. Il est urgent de remédier à une telle situation. L'ordre public et la sécurité se trouvent en effet au fondement de la vie en société et de l'exercice des libertés. Assurer la sécurité de nos concitoyens est l'une des missions les plus essentielles de l'État. Même si d'autres acteurs y concourent au sein d'un « continuum de sécurité », c'est à l'État qu'il revient de faire respecter les lois sur le territoire national et de permettre une activité sereine. Les policiers municipaux et les gardes champêtres sont un important pilier. Ces agents sont présents en permanence sur les territoires des communes qui ont pu les recruter. Ils sont proches des habitants et de leurs préoccupations. Nous soutenons donc l'expérimentation visant à confier à certaines polices municipales des prérogatives de police judiciaire. Elle permettra de déterminer le bon niveau d'exercice de ces compétences. À ce titre, nous insistons sur la nécessité d'une bonne complémentarité entre les polices nationale et municipale, notamment l'indispensable compatibilité entre leurs outils informatiques. Il faut néanmoins prendre garde à ne pas creuser davantage le fossé entre la ville et la campagne. Toutes les communes n'ont pas les moyens de recruter des agents de police municipale, et nombre de celles qui ont pu en recruter ne disposent pas d'effectifs suffisants pour participer à l'expérimentation prévue à l'article 1. Je me félicite à cet égard de ce que la commission des lois ait abaissé le seuil à quinze agents. La question de la pérennisation de l'expérimentation se posera nécessairement. Il faudra veiller à ce que les petites communes ne soient pas pénalisées à cette occasion et que la sécurité soit uniforme sur l'ensemble de notre territoire. L'autre acteur de la sécurité est le secteur privé. Nous soutenons l'encadrement de la sous-traitance, qui améliorera la clarté de l'exécution de ces contrats. Dans les domaines de l'accès à la profession et du contrôle par le Cnaps, la commission a proposé des rééquilibrages bienvenus, qui devraient emporter l'adhésion.

Les récentes décisions de la CNIL et du Conseil d'État interdisant l'usage de drones munis de caméras à des fins d'ordre public impliquaient de définir le régime légal de leur utilisation. S'il est important de donner à nos forces de l'ordre un accès à cette technologie, il est indispensable d'encadrer son usage pour protéger les libertés publiques et garantir la validité des procédures fondées sur de tels éléments de preuve. À cet égard, je me réjouis que la commission ait pris en compte les recommandations de la CNIL. L'encadrement proposé est à même de renforcer la confiance placée dans la vidéoprotection. Par ailleurs, nous soutenons le choix d'écarter la possibilité offerte aux forces de l'ordre de diffuser des images aux fins d'information du public sur les circonstances d'une intervention. Il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Enfin, concernant le renforcement de la protection des forces de l'ordre, nous regrettons que l'article 24 ait été la source de vives polémiques, alimentées par des déclarations malheureuses. Il faut défendre ceux qui nous défendent. En la matière, la rédaction proposée par nos rapporteurs nous semble meilleure, sans qu'elle parvienne toutefois à résoudre toutes les difficultés. Nos forces de l'ordre ont avant tout besoin de moyens matériels suffisants pour remplir leur mission sereinement. L'ensemble des mesures figurant dans ce texte contribue à l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens. La question des moyens financiers consacrés à nos forces de l'ordre reste cependant centrale. Nous serons à vos côtés, monsieur le ministre, chaque fois qu'il sera question d'améliorer les conditions

alors que le contexte de crise sanitaire a déjà fortement ébranlé nos libertés individuelles et collectives, le Gouvernement et la majorité LaREM font le choix de les miner plus encore

conçue à l'origine pour acter un élargissement des compétences de la police municipale, s'est vue détournée de son objet principal. Elle est en réalité pilotée par le Gouvernement, lui-même aux ordres des syndicats de police les moins progressistes, et impose des dispositions dangereuses, dénoncées par maints observateurs, dont les rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Défenseure des droits et la CNCDH. La version du texte qui nous est soumise ne saurait satisfaire mon groupe, compte tenu des nombreuses atteintes aux droits et libertés fondamentales qu'elle comporte toujours et le peu de garanties qui ont été introduites. Certaines modifications apportées par la commission des lois peuvent, bien sûr, être saluées. Celle-ci a, par exemple, supprimé l'article 20 qui prévoyait la transmission d'images provenant des systèmes de vidéoprotection installés dans les parties communes d'immeubles.

Le réel problème que soulève l'article 24 n'a cependant pas été réglé. L'infraction prévue porte encore atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression ; elle crée un obstacle supplémentaire au contrôle des policiers et des gendarmes et, par conséquent, à l'action de la justice. Steve Maia Caniço, Cédric Chouviat, Michel Zecler, nous avons tous à l'esprit ces victimes dont nous n'aurions rien su ou qui n'auraient pas pu se défendre sans ces images.

concernent le déploiement et l'intensification de la vidéosurveillance, ce à quoi nous, écologistes, nous opposons. Entre surveillance de masse « en marche » et instillation de la peur, ce gouvernement a fait le choix de la doctrine Big Brother. L'usage des drones, particulièrement intrusif, inquiète légitimement, tant il est lui aussi susceptible de brider la liberté de manifester. Nous disons également non au maintien de l'article 25, qui prévoit la possibilité, pour les policiers nationaux et les militaires de la gendarmerie, de conserver leur arme en dehors des heures de service et dans des établissements recevant du public. Reconnaissons enfin que ce texte n'a hélas de « global » que le nom. Il manque d'ambition et ne s'appuie sur aucune vision complète et réellement novatrice de la sécurité en France. Rien n'a été pensé quant à la formation des policiers, notamment sur les questions de la lutte contre tous les types de discrimination. Rien n'a été envisagé non plus pour remédier aux contrôles au faciès, aux violences policières ou encore à cette culture de l'impunité qui jette le discrédit sur l'image des forces de l'ordre, et contribue à saper le lien de confiance

Prétextant une situation sécuritaire dégradée, le Gouvernement alimente en réalité, et sans réel fondement, une surenchère sécuritaire dans notre pays au travers de ce projet de loi déguisé en proposition de loi. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera contre ce texte. Mes chers

légitime. Néanmoins, je suggère au Sénat d'observer qu'aucun des cadres classiques du droit de la sécurité publique, ces cadres éprouvés et reconnus comme constitutionnels qui sont la base de notre législation dans les trois domaines concernés, n'est affecté par les dispositions de ce texte, tel qu'il nous arrive de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un texte de moyens

un mot de diagnostic. Les effectifs disponibles sont en progression dans les trois ensembles : police et gendarmerie nationales, police municipale, y compris gardes champêtres, et sécurité privée,

ce texte lance une expérimentation de grande ampleur, ouvrant aux polices municipales comptant plus de quinze agents qualifiés la capacité de relever des infractions dans plusieurs champs qui- nous le savons tous -comptent beaucoup dans l'atmosphère de sécurité locale. J'en cite quelques-unes, pour montrer que l'on n'est pas non plus en train de bouleverser l'équilibre des pouvoirs : la vente à la sauvette, les infractions à la législation des débits de boissons et de l'ivresse publique, la dégradation de biens publics, le défaut de permis de conduire et d'assurance, les obstacles déposés sur la voie publique, l'intrusion sur les terrains communaux ou dans les locaux communaux, les occupations de parties communes d'immeuble

Bien sûr, il peut y avoir un débat, tout à fait justifié et respectable, sur certaines de ces capacités, mais le cadre me semble particulièrement sécurisant du point de vue des libertés, puisque cette évolution

à propos d'un « retrait » ou d'un « transfert » de la police nationale. Je veux le souligner devant les collègues qui ont tenu ces propos, rien, dans ce texte, ne prévoit un retrait quelconque des prérogatives de la police ou de la gendarmerie nationales, ce qui serait d'ailleurs

de sorte que le rapport entre employeur, champ géographique et type d'autorité soit bien clarifié, pour les cas, nombreux, où une communauté n'est pas en mesure d'assurer cette mission.

du code de la sécurité intérieure qui énumèrent, de façon limitative, les interventions et les droits d'action des sociétés de sécurité privées n'est modifié. Ce qui change, ce sont les règles de recrutement, de formation et de discipline, ainsi que les conditions de contrôle

La proposition de loi Fauvergue-Thourot fait tout d'abord la part belle au renforcement des pouvoirs et du rôle des polices municipales, aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie. Nous mesurons bien l'intérêt qu'a l'État,

C'est pourquoi nous avons souhaité encadrer plus encore la sous-traitance, dont la multiplication des maillons est une menace pour l'efficacité et la sûreté des missions de ces sociétés. Nous avons également entendu réaffirmer le rôle de la CNIL dans le contrôle de ces entreprises ; nous sommes prêts à doter cette autorité de régulation de moyens dédiés suffisants. De plus, le secteur de la surveillance fait appel à l'utilisation massive et sans doute croissante de la vidéoprotection. Nous avons donc voulu ajouter une obligation de moyens concernant la protection des données. J'en viens à l'article 24, réécrit par les rapporteurs de la commission des lois. En la matière, notre seule boussole est la Constitution. Il est indispensable que la police républicaine puisse accomplir son travail d'interpellation sans crainte pour la vie de ses Il est indispensable également que la liberté de la presse soit préservée, de même que notre droit commun à la sûreté, c'est-à-dire l'assurance, pour le citoyen, que le pouvoir de l'État ne s'exercera pas sur lui de façon arbitraire et excessive.

Je terminerai en évoquant le recours aux drones de surveillance. Ce sujet mériterait un autre texte, plus approprié et plus approfondi. Donc, comment pouvons-nous accepter que, en plein examen de ce texte, un décret autorise par ailleurs la surveillance à des fins statistiques du port du masque dans les transports ? Est-ce bien le moment ? Est-ce urgent, alors que la confiance dans la surveillance est si entachée ? Comme le disait Voltaire, « la modération est le trésor du sage » ... Mes chers

groupes, avons été confrontés très tôt, en tant qu'élus locaux, à ces questions. On nous a d'ailleurs parfois montrés du doigt, accusés,

Je rappelle cette évidence, parce que ce sentiment d'insécurité est d'abord un vécu lié à une violence subie et parce que ce sentiment, ce vécu, touche en premier lieu les classes populaires. Oui, monsieur le ministre,

nous l'idée de remettre en cause l'initiative parlementaire, mais, pour une mission régalienne aussi importante que la sécurité, un projet de loi eût été judicieux, afin de bénéficier, par exemple, d'une étude d'impact, avis du Conseil d'État ou de la CNIL sur des sujets majeurs tels que la légalisation des drones, la diffusion en direct des images des caméras-piétons au centre d'opérations ou encore les nouvelles prérogatives de la police municipale. la police municipale, justement, le renforcement des missions et des compétences des agents de cette force suscite des questions, car ces derniers relèvent d'un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale et ils n'ont pas la même formation que les gardiens de la paix et les gendarmes. Cette proposition de loi contribue à une confusion entre les différents corps de police, alors que les polices municipales sont sous la hiérarchie des maires et qu'il y a, de ce fait, autant de doctrines d'emploi que de communes.

L'urgence est de s'atteler au renforcement des moyens de la police nationale, dans sa mission de service public et de proximité, par le recrutement de nouveaux policiers nationaux formés à renouer le lien avec la population.

équilibre entre protection de l'ordre public et respect des libertés publiques. Le travail de réécriture de la commission des lois, parfois efficace, demeure à nos yeux bien en deçà des attentes ; nous y reviendrons au cours de la discussion des articles. à l'examen de ce texte, je dirai que penser, proposer et agir pour la sécurité, pour toute la sécurité- tant celle du quotidien, dans nos quartiers et nos communes, que celle qui permet d'assurer la protection de notre État, de notre République -, c'est tirer les conséquences des errements de la politique conduite depuis 2002, de l'abandon de la police de proximité, à l'origine des graves dysfonctionnements que nous constatons au quotidien. Penser la sécurité, c'est rétablir le lien de confiance entre les forces publiques et la population. Enfin, penser la sécurité, c'est répondre à la souffrance et aux conditions de travail extrêmement difficiles des fonctionnaires de police et de gendarmerie.

de cette inflation législative galopante ... D'ailleurs, le problème n'est sans doute pas tant dans la multiplication des textes que dans leur inefficacité relative. Je tiens à adresser aux auteurs de cette proposition de loi un message amical leur initiative législative initiale ne méritait pas forcément le tombereau de commentaires provoqué par ce texte depuis que le ministère de l'intérieur a souhaité reprendre la plume. J'en profite également pour saluer très sincèrement le travail de nos deux rapporteurs, ! ... qui ont décrit la genèse de cette proposition de loi avec force détails. Pour résumer, nous avons affaire à une proposition de loi écrite par deux députés puis modifiée par le ministre de l'intérieur, avant qu'un article problématique, l'article 24, ne devienne l'objet des convoitises de différents collectifs, différents collectifs, se caractérisant d'abord par l'irrespect de la procédure parlementaire ; on se souvient du groupe de travail ; on n'est pas loin du « séparatisme » constitutionnel a multiplié, ces dernières années, les manoeuvres de diversion. Dois-je le rappeler, ce texte arrive après un schéma national du maintien de l'ordre. Dois-je le rappeler, ce texte arrive avant un « Beauvau de la sécurité », qui démontre la non-pertinence du fameux « continuum de sécurité », puisque n'y interviennent que des représentants de la police nationale et de la gendarmerie, laissant police municipale et sécurité privée sur le pas de la porte ... Dois-je le rappeler, nous aurons, après cela, un projet de loi pluriannuelle de programmation, si nous n'avons pas, auparavant, un texte contre les bandes, un autre contre les feux d'artifice et, peut-être, si nous sommes sages, un troisième contre les islamo-gauchistes .... Le problème ne viendrait-il pas plutôt de l'incontinence législative en matière sécuritaire ? Un fait divers ? Une loi ! Un « tweet » de travers ? Une loi ! Le Conseil constitutionnel censure une loi ratée ? Tentons de la faire repasser ! Ce ras-le-bol lié à l'accumulation des lois, je l'ai entendu dans la bouche de tous mes interlocuteurs- policiers, gouvernementales (ONG) -et ce n'est pas qu'une question de forme ; c'est une question de fond. Ainsi, on nous dit qu'il existe déjà six dispositions législatives permettant de répondre aux problèmes que cherche à résoudre l'article 24 ; six ! Le Gouvernement en ajoute une autre avec cet article et

a déjà commencé à faire entendre la ligne de la chambre des territoires sur ce continuum de sécurité. Cette ligne, c'est que nous sommes quelque peu dubitatifs ... La complémentarité entre police nationale et police municipale est un objectif louable,

Comment organiser un continuum, quand il n'y a pas de continuité, puisqu'il n'existe pas de police municipale partout et que cette police n'a pas, partout, les mêmes objectifs ni les mêmes moyens ? Comment assurer la continuité, quand certaines collectivités, plus riches et plus attrayantes, attireront mécaniquement le gros des groupes ? Le continuum de sécurité signifie-t-il que la police municipale de ma commune doit être considérée comme une force antiterroriste ou comme une police de la tranquillité et de la proximité ? Les responsabilités des policiers municipaux et celles des policiers nationaux se recoupent-elles ? Leurs membres sont-ils contrôlés de la même manière ?

L'encadrement de la sécurité privée, recherché au travers de ce texte, représente un objectif louable. Les forces de sécurité privée constituent une composante non négligeable de la sécurité dans notre pays. l'on s'en félicite ou non, c'est quelque chose de dorénavant ancré relativement profondément dans notre pays et il est bienvenu d'essayer d'améliorer les choses en la matière. Une réforme plus forte du Cnaps aurait sans doute été préférable et l'on pourra discuter des mesures précises en la matière, mais, sur la philosophie, nous sommes d'accord. J'aborde maintenant ce qui constitue le troisième axe de ce texte : la question des images, seule solution trouvée pour aborder les rapports entre police et population dans ce texte. On sait la frilosité traditionnelle du ministère en la matière : les citoyens et associations engagés n'ont ainsi pas été invités au Beauvau de la sécurité. Les caméras-piétons ne font pas disparaître les tensions entre la police et la population ; elles les documentent. C'est d'ailleurs la même chose pour tout dispositif de captation vidéo : ce ne sont jamais des solutions miracles ; ce sont toujours des outils, non des fins en soi. Comme ce sont des outils, il faut en assurer une utilisation saine. Je salue d'ailleurs le travail de Loïc Hervé, dont la qualité de membre du collège de la CNIL a sans doute permis d'écrire des amendements souvent bienvenus. Sont-ils suffisants ? À gauche, nous en doutons. Vous l'aurez compris, nous abordons l'examen de ce texte en étant critiques mais ouverts sur les améliorations que notre chambre pourra apporter. Cette loi de « sécurité bancale » n'appelle ni enthousiasme ni construction de barricades. Elle exige d'abord notre vigilance et notre travail, au cours de cette semaine d'examen. Police nationale, forces de sécurité privées, gardes champêtres, avocats, magistrats, citoyens engagés ; tous n'ont pas la même vision du monde, mais nous devons partir du principe qu'ils sont tous dans le même camp, pour reprendre, en les retournant, les propos d'un célèbre préfet. La sécurité c'est l'affaire de tous, policiers avec citoyens, gendarmes avec juges, municipaux avec avocats et j'irais même jusqu'à dire : majorité avec oppositions ! La balle est donc dans votre camp, monsieur le ministre. Puisque,

Notre commission l'a bien amendé ; elle en a même réécrit certains articles, comme l'article 24. Elle contribue ainsi à tirer le Gouvernement d'un mauvais pas. Le Sénat reprend à son compte l'exigence d'une protection accrue des policiers et des gendarmes, tout en préservant intégralement la liberté des journalistes. Je remercie notre rapporteur, Marc-Philippe Daubresse, d'avoir su imaginer une solution très pertinente

que nul n'est besoin de nommer une commission gouvernementale pour corriger un texte adopté par l'Assemblée nationale. Chaque assemblée est là, précisément, pour affiner le travail législatif de l'autre. Il serait temps de réfléchir à une méthode de prévention des accidents législatifs, qui paraissent se multiplier en cette fin de quinquennat ... On reproche parfois au Parlement de ralentir le travail gouvernemental, mais on pourrait tout aussi bien reprocher au Gouvernement sa boulimie législative, M. Durain vient de le dire. Il semble que les gouvernements s'ingénient de plus en plus à faire passer leurs projets des propositions de loi. Il suffit alors de mettre en oeuvre la procédure accélérée et le tour est joué. La semaine d'initiative parlementaire, voulue par Nicolas Sarkozy, redevient gouvernementale ; le texte peut alors aboutir dans des délais records, sans étude d'impact, sans consultation du Conseil d'État ni de la CNIL, sans délibération du conseil des ministres et avec une inscription ultrarapide à l'ordre du jour. L'abcès de fixation de l'article 24 démontre que ce détournement de procédure a ses limites ; l'improvisation législative se paye comptant. Je tiens aussi à saluer l'initiative prise par le président Buffet, qui a consulté la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis de celle-ci s'est révélé précieux et notre rapporteur Loïc Hervé s'en est fortement inspiré. La volonté de renforcer l'utilisation des technologies de sécurité ne peut pas aboutir au détriment des libertés, c'est évident. Tel qu'il a été amendé par notre commission, le texte dont nous sommes saisis présente un réel intérêt pour la sécurité publique. L'aggravation continue de la violence au cours des années récentes, la multiplication des agressions et des actes de vandalisme en marge des manifestations, les violences toujours plus grandes en opposition à l'action des forces de sécurité, ajoutées à la mobilisation intensive de notre appareil de sécurité pour faire face à la menace terroriste, mettent à rude épreuve policiers et gendarmes. L'inversion des réalités est à l'oeuvre à travers les mises en cause à répétition du recours à la force légale. C'est une manière insidieuse, dans certaines travées, de transformer les défenseurs de la loi en agresseurs et les agresseurs en victimes. Faut-il le rappeler, l'usage régulier de la force au nom de la loi ne constitue pas une violence ; le recours à la contrainte légale est même une des raisons d'être de la police et de la gendarmerie. Si tout abus dans l'exercice de la contrainte légale doit être sanctionné, il faut, tout de même, avoir le courage de dire que les violences policières demeurent heureusement très rares, tandis que les violences dont sont victimes les représentants des forces de sécurité sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, le nombre d'agressions contre des gendarmes a augmenté de 76 % en dix ans plus de 10 000 policiers et gendarmes sont blessés en mission chaque année. La première condition de la sécurité des Français est donc bien la protection des agents des forces de l'ordre et le renforcement de leurs moyens d'action. Nous n'allons pas reprocher au Gouvernement de s'en préoccuper enfin ; il serait même bien inspiré de s'en tenir désormais à cette ligne claire, en rompant avec l'ambiguïté du « en même temps » qui était encore à l'oeuvre ces derniers mois, quand certaines méthodes d'interpellation ont brusquement été interdites pour éteindre une polémique venue d'Amérique, avant même que de nouvelles méthodes aient pu être enseignées aux policiers. Les travaux de nos collègues Catherine Di Folco et Maryse Carrère ne manqueront pas d'éclairer notre assemblée sur ces questions. Pour autant, le Sénat, fidèle à sa vocation de défenseur des libertés, doit aussi être attentif à ce que les moyens des forces de sécurité soient strictement proportionnés aux objectifs qui leur sont assignés. Ainsi l'exploitation d'images de vidéosurveillance ou de caméras-piétons sera-t-elle strictement encadrée- merci, monsieur Hervé ! Quant aux drones, ils doivent pouvoir être utilisés, par exemple, pour contrôler des mouvements de rue, pour suivre des commandos de Black Blocs- il y en a ! -, pour empêcher des actes de vandalisme, mais il est impératif que le dispositif législatif retenu garantisse la protection de la vie privée. Enfin, les dispositions relatives à la police municipale devraient permettre un meilleur continuum entre police locale et police nationale, mais sans faire peser sur les maires des responsabilités qui ne peuvent relever que de l'État, lequel ne saurait se défausser sur eux. Comme l'a montré Marc-Philippe Daubresse, la bonne articulation des missions des uns et des autres sera gage d'efficacité. Pour toutes ces raisons, les propositions de notre commission en vue d'améliorer ce texte utile, bien que mal né, me semblent devoir être approuvées par le Sénat.

l'excellent travail de nos rapporteurs, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, l'écoute et la rigueur dont ils ont fait preuve pour ce texte quelque peu délicat, dont le contexte et les conséquences nous invitent à dépasser frénésie et posture. Le Sénat a aujourd'hui la responsabilité d'oeuvrer à la recherche de l'équilibre entre libertés individuelles et sécurité, socle du contrat social qui fonde notre démocratie. La cohabitation de ce texte avec d'autres initiatives, telles que le Livre blanc de la sécurité intérieure, le Schéma national du maintien de l'ordre ou le Beauvau de la sécurité, atteste de la nécessité, mais aussi de la difficulté, d'adapter la loi aux évolutions de la délinquance et de la violence, ainsi qu'à celles des technologies, peuvent permettre, par l'image, de transformer parfois si douloureusement ceux qui nous protègent en cibles et en victimes tragiques. Cette violence, qui va de l'incivilité à la délinquance, à l'agression, à l'attentat, se répartit tristement, mais certainement, dans tout le territoire et gangrène notre cohésion sociale. Nos rapporteurs, et la commission des lois, monsieur le président Buffet,

Le Sénat l'a en quelque sorte ciselé, en relevant le défi de renforcer la sécurité, de mieux protéger la police, de préserver la liberté de la presse et la nécessaire transparence envers les citoyens.

Les images captées par la police doivent garder un caractère exclusivement probatoire et non participer à l'alimentation des directs des chaînes d'info.

en dehors des heures de service dans un établissement recevant du public ? Quand l'actualité s'efface, et avec elle l'émotion qu'elle a suscitée, la menace reste, elle,

lequel ne saurait la transférer aux collectivités ou la diluer. Seule la tranquillité du voisinage peut relever de la police du maire. La création d'une police municipale et son dimensionnement relèvent de la seule et libre initiative des conseils municipaux, mais force est de constater la montée en puissance de la police municipale, par nécessité très souvent, pour gérer plus efficacement les incivilités du quotidien et, parfois, pour pallier la carence de l'État dans certains domaines. Ensuite, l'expérimentation proposée sera, et devra rester, volontaire, à l'initiative des communes, comme devra l'être son élargissement éventuel à l'issue de la période d'expérimentation.

une évaluation précise et transparente. Si toute expérimentation nécessite une évaluation, celle-ci s'impose pour cette disposition à deux titres : parce qu'il s'agit d'une compétence régalienne, mais

en réaffirmant que la sécurité est un pilier de la démocratie, mais qu'il faut tout autant protéger les libertés, ce que la sécurité doit permettre de faire. Notre pays est secoué par un sentiment d'insécurité croissant, qui ne peut être ignoré ou méprisé. Il faut nommer les choses pour les endiguer, car la peur est très mauvaise conseillère. S'il n'y a pas de liberté sans sécurité, la sanction, monsieur le ministre, est, au mieux, curative et ne saurait suffire à guérir nos maux sans une mobilisation collective de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi de la famille en faveur de l'éducation, de la prévention et de l'intégration, sans la juste efficience et réactivité de la justice. J'ai bien compris que ce volet fera l'objet d'un second épisode, qui interviendra très prochainement avec le garde des sceaux. Comme il faut un village pour aider un enfant à grandir, c'est la Nation tout entière qui doit se mobiliser pour endiguer ce fléau, mais aussi pour protéger ceux qui protègent la République et nous protègent, et dont nous devons saluer l'engagement, qu'ils payent parfois de leur vie. La parole

ainsi va le monde et vous ne changerez pas le devenir de la société en limitant le nombre de lois ! On bouge, tout bouge. La définition de la sécurité n'est pas la même aujourd'hui que celle qui prévalait avec un Sartine sous Louis XV, un Fouché sous Napoléon Iou un Persigny sous Napoléon III. À l'époque, la sécurité relevait d'un maillage au profit du régime.

de soutien, de pilier de la République. Ce sont devenus deux éléments clés, fondateurs, permanents, de la possibilité pour la République de se défendre

opinion politique. J'admets très bien, madame Assassi, que tous les rangs, tous les camps et tous les groupes politiques peuvent soutenir la police et la gendarmerie.

Il faut renverser la charge de l'inquiétude : il faut que les citoyens qui vivent normalement dans un cadre légal

La même commission est saisie au fond pour deux textes consécutifs, ce qui représente une charge de travail extrêmement lourde pour tout le monde : les parlementaires, leurs équipes, les groupes et l'administration. Cela nuit à la qualité du travail législatif, dont le Sénat se fait pourtant une fierté. De surcroît, nos débats vont se croiser, puisque nous examinerons le fameux article 24 en séance et, parallèlement, en commission, l'article 18 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, tous deux relatifs à la diffusion d'informations ou d'images concernant les dépositaires de l'autorité publique. Nous comprenons que le Gouvernement souhaite tenir son agenda chargé avant la fin du quinquennat, mais cela ne peut se faire au détriment de la qualité du travail parlementaire. Je souhaite donc attirer votre attention, madame la présidente, mes chers collègues, sur la nécessité de garantir cette qualité. Acte vous est donné de ce

un encadrement plus rigoureux de l'expérimentation des nouvelles attributions judiciaires des agents de police municipale. Cet encadrement correspond aux recommandations qui figurent dans le rapport que j'ai réalisé avec notre collègue Corinne Féret, relatif l'ancrage territorial de la sécurité intérieure et qui a été présenté le 28 janvier dernier devant la délégation aux collectivités territoriales. Dans le cadre de nos travaux, nous avons été témoins des préoccupations des élus locaux. Les maires sont soucieux de contribuer à l'émergence d'un véritable continuum de sécurité, mais ne veulent pas servir de palliatif au désengagement de l'État.

Les amendements adoptés en commission à l'article 1 réduisent le risque de voir peser sur les communes, à terme, de nouvelles charges non compensées, au mépris de l'article 72-2 de la Constitution. Ainsi cet article 1 partage-t-il l'esprit de notre rapport, lequel appelait à accepter avec vigilance l'expérimentation des nouvelles compétences des polices municipales. Les maires doivent rester libres

Aussi, et conformément à l'une des conclusions de ce travail, il nous semble qu'il convient de préciser le champ de l'évaluation intermédiaire prévue par la commission des lois du Sénat.

ils sont donc contraints de rédiger leurs écrits sur papier, ce qui ralentit le traitement procédural et engorge les services judiciaires, sans compter que le montant des contraventions n'est souvent pas dissuasif. En 2011, la Cour des comptes indiquait que les polices municipales étaient souvent plus présentes sur le terrain que la police nationale, sans pour autant opposer les unes à l'autre.

impact réel sur les services de l'officier du ministère public. Par ailleurs, les infractions aux arrêtés du maire- contraventions de première classe, jusqu'à 38 euros -ne sont pas forfaitisées. Elles nécessitent donc, là aussi, un traitement lourd et coûteux, alors même qu'elles représentent une grande partie de l'activité contraventionnelle. La faiblesse du montant des amendes, l'absence de dématérialisation et de forfaitisation génèrent donc beaucoup de déchet, ce qui obère en même temps l'action publique et les politiques locales de sécurité conduites par les maires. Les possibilités procédurales n'étant pas en adéquation avec l'impact humain de la police municipale, il paraît important de modifier l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, en le complétant de la liste des infractions actuellement relevées par les agents de police municipale, méritent une amende forfaitisée. Monsieur le ministre, les maires sont en attente des arrêtés que vous pourriez prendre en ce sens. La parole est à Mme Cécile Cukierman,

de nombreux courriers d'élus locaux, de parlementaires, qui vous ont alerté sur la baisse des effectifs. Les deux dernières lois de finances ont introduit quelques corrections en ce sens, mais vous savez comme nous que les effectifs sont encore insuffisants dans nombre de nos commissariats pour répondre à cette problématique du quotidien et à ce ras-le-bol que vivent

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'illusion que l'État central est capable de prendre en charge toutes les facettes de la sécurité s'est largement dissipée, y compris dans l'esprit de nos concitoyens. Nous ne discutons pas ici de la création de la police municipale : elle existe

Nous assumons que l'État délègue à des acteurs locaux la gestion de tâches relevant de l'idée de proximité, mais je voudrais citer à mon tour le rapport de Corinne [L']extension de la compétence de la police municipale peut être perçue par certains élus locaux comme une forme de désengagement de l'État, alors que la sécurité est une mission régalienne qui lui incombe prioritairement. » Je ne peux que saluer cette conclusion. Nous souhaitons, mes chers collègues, que les polices municipales soient des partenaires fiables de nos forces de l'ordre. Élargir leur champ d'intervention n'apparaît pas d'emblée comme une mauvaise chose, je vous le concède, mais nous souhaitons plus de garanties sur l'encadrement de cette extension ; nous demandons que soit mis en place un contrôle, celui de la commission consultative des polices municipales, condition condition pour maintenir un lien de confiance entre la population et sa police municipale. Nous souhaitons également que le champ des actions déléguées relève bien de l'action de proximité. C'est pourquoi l'extension des pouvoirs de la police municipale doit être circonscrite aux actions qui relèvent traditionnellement de la police de la

La CNCDH déplore, [ ...], l'attribution croissante de missions de police judiciaire à la police municipale. Cette tendance ne va pas dans le sens d'une pacification des rapports entre la police et la population, et ne peut qu'encourager un désengagement de l'État et de la police nationale au profit d'agents chargés de mettre en oeuvre les priorités de certains élus locaux, particulièrement sensibles aux enjeux électoraux.

Les polices municipales doivent assurer la tranquillité publique au sein de nos territoires ; elles sont des agents du vivre ensemble. Elles doivent apaiser l'espace commun et, donc, acquérir la confiance des habitantes et des habitants. Tel est le coeur de leurs missions, dont on commence un peu à les détourner.

Vous prévoyez que les polices municipales soient chargées, par voie d'expérimentation, de plusieurs missions normalement dévolues à la police nationale. Alors qu'au niveau local nous devons privilégier une approche globale, multisectorielle et non uniquement centrée sur la répression,

l'insécurité, d'autre part : ces facteurs poussent un certain nombre de personnes à commettre des actes délictueux en lien avec le chômage, la misère, la non-éducation et, parfois, la mauvaise intégration sur le territoire national,

En l'espèce, l'article 1 octroie des compétences de police judiciaire à la police municipale. Du fait de l'inégalité de ressources entre les communes, cette délégation de compétences pourrait conduire à des inégalités de traitement entre les citoyens et à un morcellement de l'action des forces de l'ordre sur le territoire. Surtout, deux visions de la police municipale en France s'opposent. Il y a la vision classique, celle que mon groupe et moi-même portons : une police de proximité qui met l'accent sur la prévention et la gestion des conflits ainsi que sur l'accueil et la prise en charge des victimes et la protection des populations les plus vulnérables. Cette police offrirait en particulier des services de proximité aux femmes et aux enfants victimes de violences de violences ; non équipée d'armement létal, elle ferait même de la très grande proximité au contact des habitants, des associations, des commerçants, etc. Elle serait notamment formée aux luttes contre les discriminations et et serait, par sa mixité et sa parité, à l'image des citoyens qu'elle accompagne et protège au quotidien. Il y a la vision que proposent les ce texte : une police municipale dont les missions ressemblent à celles d'une police nationale- prétendu continuum de sécurité, en réalité symbole d'une confusion de compétences entre les différentes forces de sécurité, à laquelle

Cet article transfère des compétences de police judiciaire aujourd'hui exercées par des policiers nationaux et par des gendarmes à des policiers municipaux, sous certaines conditions de taille et d'organisation de service. de service. Il convient de rappeler que la police municipale est placée sous l'autorité du maire, alors que les forces de sécurité de l'État agissent sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire.

Il conduit par ailleurs à une situation d'insécurité juridique. On assiste là à un glissement d'une police de la tranquillité, de la médiation, de la prévention, une police locale, vers une police de sécurité, l'État se déchargeant au passage de ses responsabilités sur les communes qui devront, pour les assumer, sortir leur portefeuille. L'État doit garder tout ce qui est du domaine régalien et du champ judiciaire. Le continuum républicain de sécurité doit garantir la cohérence de l'action publique et lutter contre les disparités locales. Or cette expérimentation crée un continuum à plusieurs vitesses, selon que l'on est volontaire ou non pour l'expérimentation, selon que l'on en a ou non les moyens, selon que l'on est une grande ville ou un village. La sécurité efficace, monsieur le ministre, c'est celle qui est exercée par une police républicaine retrouvant le lien avec les Français, une police et une gendarmerie dotées des moyens nécessaires, de principes déontologiques clairs et de temps de formation suffisants. La République est une et indivisible. À ce titre, elle doit garantir un égal accès à la sécurité à tous les citoyens sur l'ensemble du territoire. L'article 1, en introduisant cette expérimentation et ce transfert de compétences de police judiciaire, remet en cause ce principe. C'est la raison pour laquelle je demande à mon tour sa suppression.

Dans le texte proposé, les rapporteurs ont pris soin d'être très exigeants sur l'évaluation et- nous le verrons certainement tout à l'heure -sur l'atterrissage de l'expérimentation, pour éviter un élargissement.

tout en réaffirmant que la sécurité est une compétence régalienne et qu'il ne s'agit nullement d'un transfert déguisé, mais d'une meilleure réactivité demandée par certains élus. La parole

la différenciation en dehors des lois de la République et de l'unicité de celle-ci ! Reconnaître la différence et la spécificité ne veut pas dire remettre en cause les règles de la République.

peut-on répondre au besoin de République partout dans notre pays

tout en veillant, dans le cadre d'un protocole négocié avec le préfet, à ce que les responsabilités des uns et des autres soient clairement déterminées.

a été supprimée et que ces policiers manquent dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos villages. Il ne faut pas déplacer le problème ! Donner aux polices municipales la possibilité d'exercer des compétences de police judiciaire, c'est un vrai problème.

M. Alain Marc. L'exercice de la police administrative générale est une prérogative historique du maire. Toutefois, les débats à l'Assemblée nationale sur l'expérimentation créée à l'article 1 de cette proposition de loi ont pu laisser penser que la création d'un SIVU chargé du fonctionnement des policiers intercommunaux reviendrait en réalité à lui déléguer le pouvoir de police. Cet amendement tend à affirmer dans la loi que la mise en place d'une telle expérimentation n'est pas de nature à remettre en question l'exercice du pouvoir de police par le maire.

Toutefois ce seuil demeure trop élevé. Il pénalise les communes de petite taille, souvent situées en milieu rural et hyper-rural. Si l'objet de la proposition de loi est de permettre aux collectivités locales d'accompagner l'État dans son devoir d'assurer la sécurité en veillant, notamment, sur l'ensemble du territoire de la République au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens, cela ne peut se faire au seul bénéfice des grandes agglomérations urbaines. La problématique de la délinquance au quotidien touche

parole est à M. Alain Marc. L'augmentation de l'insécurité concerne malheureusement l'ensemble du territoire, et pas seulement les grandes villes. Dans les faits, le seuil de vingt agents ne correspond pas à la répartition des effectifs des polices municipales sur le territoire national, puisque la moyenne nationale révèle un effectif moyen de 4,9 agents pour 10 000 habitants. Imposer un tel seuil revient également à méconnaître le fait que nombre de ces services ne comptent ni directeur de police municipale ni chef de service de police municipale, mais sont pourtant commandés par un brigadier-chef principal.

existants. Le présent amendement vise à adapter à la réalité et à la diversité de nos territoires les conditions de seuil et d'encadrement de l'expérimentation. Ainsi, il tend à laisser la possibilité à l'ensemble des communes ayant au moins trois agents de police municipale, dont un brigadier-chef principal,

Mme Laurence Harribey. L'article 1 permet, par dérogation aux règles du code de procédure pénale qui prévoient une transmission par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire aux agents de police municipale d'adresser directement leurs rapports et PV simultanément au maire et, par l'intermédiaire des directeurs ou des chefs de service de police municipale, au procureur de la République. officiers de police judiciaire étant simplement informés sans délai de cette transmission, ils ne joueront plus le rôle de filtre de la qualité et de l'opportunité de ces actes. Cette nouvelle situation, même appliquée à titre expérimental,

en particulier dans les communes les plus importantes, et nécessitera la mise en oeuvre de nouveaux cadres de partenariat entre le procureur de la République et la police municipale, conséquences auxquelles la présente proposition de loi n'apporte pas de réponse concrète. concrète. L'absence de projection de cette mesure, alors que la France est le pays en Europe qui compte le moins de procureurs par habitant et où les parquets exercent le plus grand nombre de missions, la rend inadéquate. L'amendement

Deuxièmement, la législation actuelle autorise déjà les gardes champêtres à constater les infractions et à dresser des procès-verbaux. Troisièmement, beaucoup de communes rurales et de petites communes ne disposent pas d'une police municipale. Elles sont dépendantes de la disponibilité de la gendarmerie nationale, disponibilité qui est parfois aléatoire.

dans le cadre de cette expérimentation, les gardes champêtres sont placés sous l'autorité du directeur ou du chef de service de police municipale. Il n'est donc pas utile d'attribuer cette prérogative directement aux gardes champêtres alors que le directeur ou le chef de service de police municipale bénéficiera de cette compétence.

ces amendements me renforcent dans ma conviction que cette expérimentation posera problème. Nos collègues sont déjà quasiment dans la généralisation. Abaisser le seuil de l'expérimentation,

Il ne s'agit pas de généraliser cette expérimentation à toute la France. Il s'agira au bout de l'expérimentation d'en faire le bilan et de déterminer si l'on peut continuer à professionnaliser et à renforcer la coordination entre la police nationale et la gendarmerie, d'une part, et la police municipale, d'autre part.

Je vous propose, mes chers collègues, une modification de termes dont les conséquences ne sont pas sans importance. Face à l'augmentation plus qu'alarmante du phénomène d'insécurité, l'évolution des prérogatives de nos polices municipales doit pouvoir être garantie si le maire juge que la situation dans sa commune l'exige. L'efficacité passant d'abord par la réactivité, c'est au maire, élu de terrain par excellence, de décider si les agents de police municipale ou gardes champêtres doivent exercer des compétences de police judiciaire dans le cadre de la nouvelle expérimentation prévue par cet article.

dans le respect de leurs libertés et du principe de subsidiarité auquel je suis, comme vous, mes chers collègues, très attaché, car ils sont le garant d'une démocratie incarnée, d'une action de sécurité de proximité et d'une politique publique cohérente avec la réalité des situations Cet amendement vise à réaffirmer les pouvoirs de police générale du maire et à réinstaurer l'autorité à l'échelon le plus proche des situations de conflit. Si nous voulons que la peur change de camp, il faut montrer que nos collectivités ont une force de frappe puissante, élargie et déterminée. Pour porter de nouvelles ambitions en matière de sécurité adaptées à notre présent et afin de ne pas nous laisser déborder par un futur plus violent encore, il faut leur donner une incarnation territoriale. Le maire est le premier concerné par la sécurité sur son territoire, car il est celui qui est sollicité en permanence. Il doit, dès lors, pouvoir obtenir ces nouvelles compétences de police judiciaire pour ses agents. Il n'y a pas de sécurité globale sans sécurité locale. En soutien effectif

national. Cet amendement vise à transformer une expérimentation verticale en un réel outil de coconstruction avec les territoires. Quel

pour toute infraction constatée par les policiers municipaux, qu'il s'agisse de contraventions, de délits ou de crimes. Le VI de l'article 1 de la proposition de loi prévoit d'ores et déjà une dérogation. Il ne s'agit cependant, en vertu du I de l'article 1,

La rédaction proposée supprime le caractère expérimental de la possibilité d'établir des relevés d'identité pour les délits que les policiers municipaux sont autorisés à constater.

les épisodes précédents. Nous proposons de supprimer un certain nombre d'alinéas qui visent à étendre les compétences transférées aux polices municipales dans le cadre de l'expérimentation.

a été cosigné par 58 de nos collègues. Dans l'exercice de leurs missions de sécurité du quotidien, les polices municipales sont amenées à constater des infractions ne relevant pas de leur champ de compétence. Elles peuvent ainsi être confrontées, sans le savoir, à des individus dangereux figurant sur des fichiers dédiés aux individus recherchés, violents ou terroristes, par exemple.

Il est proposé de mettre fin à cette incohérence, qui met en danger, à la fois, les agents de police judiciaire adjoints, mais également les officiers de police judiciaire lorsque leur est présenté un individu dont le caractère dangereux n'est pas encore révélé. Cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale de relever l'identité, sous l'ordre et la responsabilité de l'OPJ territorialement compétent, dès lors qu'ils sont confrontés dans le cadre de leurs interventions à une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne relevant pas de leurs prérogatives. Ce relevé d'identité ne s'inscrit pas dans le cadre d'une enquête,

vise à inscrire de manière durable dans la loi que les policiers municipaux peuvent relever l'identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater.

pour explication de vote. Monsieur le ministre, dans votre réponse à Jérôme Durain, vous tentez d'opposer les élus vertueux, qui seraient favorables aux politiques de sécurité, et les autres, qui ne feraient pas ce choix

les marges de manoeuvre des collectivités sont particulièrement restreintes aujourd'hui, et le dernier avatar qu'est la suppression de la taxe d'habitation ne va pas nous aider, particulièrement dans ce domaine.

et que les polices municipales doivent se consacrer à des missions de police de tranquillité. Cela n'empêche pas bon nombre de communes, y compris parmi celles que nous dirigeons, de consacrer de gros moyens

vous refusez que ceux qui sont souvent en première ligne, c'est-à-dire les policiers municipaux, dans le cadre d'une expérimentation et avec l'accord de l'officier de police judiciaire- aient la possibilité de simplement vérifier l'identité des individus dangereux qu'ils ont face à eux. Les policiers municipaux ne sont pas des sous-acteurs de la sécurité. En refusant de faire évoluer cet article, on les met en danger, et je le regrette.

? De la police judiciaire, du renseignement, du maintien de l'ordre ? Que restera-t-il du lien entre la police et la population ? Caricature ! Qu'est-ce que la police de la République, une fois que l'essentiel des compétences qui font la vie de tous les jours, comme vous dites, sont transférées au bloc local ?

Si nous pouvons admettre le principe d'une telle expérience, y compris au niveau intercommunal, il nous paraît essentiel que les intercommunalités susceptibles d'y participer proposent un service de police efficace. Or nous constatons que, dans certaines intercommunalités, le périmètre géographique qu'elle recouvre ne permet pas d'atteindre cette efficacité. Aussi cet amendement vise-t-il à rappeler que la taille de certains EPCI peut être un frein à une intervention équitable des forces de sécurité sur l'ensemble du périmètre retenu. Il s'agit de faire valoir la nécessité de prendre en compte dans l'organisation retenue non seulement les moyens mis en oeuvre, mais aussi leur répartition et leur capacité d'intervention mobile sur tout le périmètre concerné, et ce dans la plupart des circonstances climatiques. Si j'ai bien compris, il propose que l'arrêté ministériel qui fixe la liste des communes et EPCI participant à l'expérimentation détermine également la mise en oeuvre de cette dernière au regard de la capacité des agents de police municipale à intervenir dans un délai raisonnable sur le périmètre concerné. La mise en oeuvre effective de l'expérimentation, je l'ai expliqué précédemment, est définie localement, au cas par cas. C'est bien le maire ou l'EPCI qui est la force motrice dans les conventions de coordination. On ne va pas recentraliser par un arrêté ce que l'on doit faire sur le terrain ! C'est au maire, sur place, avec les autorités de la police nationale et de la gendarmerie, de prévoir dans une convention de coordination les modalités ainsi que les moyens au regard du périmètre concerné.

Sur ce terrain local du respect de la déontologie et de l'action des forces de police, y compris municipales, nous avons besoin, je crois, de ce type de garanties.

Deuxièmement, je m'inscris en faux contre vos propos, madame Taillé-Polian. Un arrêt de la Cour de cassation interdit aux maires d'intervenir dans l'exercice des prérogatives de police judiciaire dès lors que l'agent de police municipale est sous l'autorité fonctionnelle du procureur.

qui ne nous paraît garantir ni la sécurité des citoyens ni le bien-être des policiers et des gendarmes en France.

d'une vigilance particulière. Un déontologue peut être utile. C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

que vous devriez être également le ministre de celles et de ceux qui sont blessés, mutilés, éborgnés, tabassés par la police et la gendarmerie

Le texte initial fixe une durée de formation d'un an, alors que l'expérimentation durera cinq ans. Cette durée nous semble trop courte. À l'heure actuelle, la formation des agents municipaux est d'ores et déjà un sujet d'inquiétude pour les acteurs de terrain. Lors des auditions que nous avons menées, plusieurs magistrats et avocats nous ont alertés sur la méconnaissance de certaines procédures, qui fragilise parfois l'enquête tout entière. Nous le savons, la première constatation sur le terrain est souvent le point de départ de la procédure. Si celle-ci présente des vices de forme, c'est tout l'édifice qui peut s'écrouler. de telles difficultés existent déjà aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain quand les compétences prévues à l'article 1 seront bel et bien transférées au niveau municipal ? La formation doit être exercée tout au long de l'expérimentation : tel est le sens de cet amendement. Par ailleurs, nous souhaiterions qu'elle soit à la charge de l'État et non des collectivités.

Je ne voudrais pas qu'on sorte de cet hémicycle en pensant que les policiers municipaux reçoivent une formation bâclée prodiguée par des incompétents. Encore une fois, je veux saluer le travail remarquable effectué par le CNPFT.

J'ai bien compris que tant M. le rapporteur que M. le ministre étaient favorables à l'extension de la formation. Je voudrais vraiment insister sur la nécessité de dispenser cette formation le plus rapidement possible à compter de l'application du texte. Pour avoir été, je l'ai dit précédemment, maire d'une commune

En effet, à l'alinéa 5, l'article 1 de la proposition de loi prévoit qu'un décret déterminera les obligations de formation complémentaire s'imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres s'inscrivant dans cette expérience. Toutefois, nous voulons faire remarquer que le coût de formation constitue une charge supplémentaire pour les petites communes et les petits EPCI, et ce d'autant plus que des frais de tenue et de signalisation sont prévus également pour les gardes champêtres. Aussi, il paraît nécessaire que le décret prévoie également les modalités de prise en charge de ces frais de formation.

grâce au recours à des procès-verbaux électroniques pour l'ensemble des verbalisations liées aux compétences détenues soit par des policiers municipaux, soit par des gardes champêtres.

me semble être un gage d'efficacité, de rapidité et d'équité en condensant les procédures. Force est de reconnaître que l'établissement d'une contravention papier comporte plusieurs inconvénients, qui conduisent souvent au non-recouvrement des sommes devant être versées, notamment en raison de la longueur des procédures. Cela peut saper l'autorité du maire et contribuer à nourrir un sentiment d'impunité. D'où l'intérêt de pouvoir extraire les agents d'une logique de liste propre aux procès-verbaux écrits

De fait, la grande majorité des infractions qui sont concernées par l'expérimentation font déjà l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. Le procès-verbal électronique, qui remplace le procès-verbal manuscrit pour les infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, est déjà possible. Les policiers et gendarmes sont dotés des équipements pour faire les procédures électroniques, mais également les policiers municipaux dont la commune a décidé d'adopter ce système.

des équipes municipales candidates à cette expérimentation. Le PVE doit pouvoir être appliqué partout, tout le temps. Vous avez vous-même, madame la sénatrice Gatel, évoqué les gardes champêtres. C'est une mesure réglementaire que nous prendrons- je m'y engage. Je vais essayer de le faire d'ici à la fin de cette année. La grande difficulté que nous rencontrons, c'est que nous devons toiletter l'ensemble des amendes pour voir lesquelles peuvent être éligibles au PVE, ce qu'avait déjà fait le ministère de l'intérieur pour ses propres amendes. Vous le savez, la police nationale n'a pas encore généralisé

maintenu ? Eu égard à l'appel que nous avons lancé, aux réponses que nous avons reçues, à la confiance que nous entretenons à l'égard du rapporteur et du ministre ainsi qu'à la mission de contrôle que nous exercerons tous ensemble, je retire cet amendement.

les choses. Nous proposons la mise en oeuvre d'un mécanisme de contrôle de l'action des agents de police municipale, qui serait exercé par la commission consultative des polices municipales (CCPM). Les modalités de ce contrôle seraient définies par décret pris en Conseil d'État.

intérieure présenté au nom de la délégation aux collectivités territoriales. Ces derniers constataient l'insuffisance du contrôle dont la responsabilité repose,, sur le pouvoir hiérarchique exercé par les maires, ce qui est insuffisant au regard de l'extension du champ d'intervention des polices municipales ainsi que de la banalisation de leur armement. Nous proposons d'aller plus loin en prenant en compte la question du contrôle mené par le ministère de l'intérieur, uniquement dans le cadre de l'évaluation de l'expérimentation. Ensuite, poursuivre la démarche de la commission des lois concernant l'article 6 B pour faire évoluer le rôle de la CCPM, afin qu'elle puisse se mobiliser sur un autre thème qui nous apparaît majeur. Sur ce sujet décisif du contrôle, le rôle de la CCPM et l'expertise de ses membres doivent être valorisés. Il est en effet nécessaire de tirer toutes les conséquences de l'orientation que va imprimer la proposition de loi sur les polices municipales avec l'extension des pouvoirs judiciaires. Enfin, le présent amendement répond à l'exigence générale d'un contrôle accru et indépendant de toutes les forces de sécurité qui est, aujourd'hui, l'une des conditions de restauration du lien de confiance entre la population et les policiers,

dans l'approche de la sécurité intérieure de notre République, notamment par le renforcement d'une police municipale rattachée à une collectivité contre une police nationale républicaine qui s'efface du fait du manque de moyens qu'on lui attribue. Cette évolution risque bien de créer un effet de cliquet qui nous empêchera de revenir sur le délitement de cette police nationale. Nous pensons donc que le Parlement doit pouvoir démocratiquement juger d'une telle expérimentation et décider d'un déploiement au niveau national, au regard des évaluations

Le Sénat étant traditionnellement opposé aux rapports, je conserve la jurisprudence défavorable.

Le dispositif proposé n'élude pas cette question en prévoyant notamment que, neuf mois au plus tard avant le terme de l'expérimentation, les communes et établissements publics concernés devront remettre au Gouvernement un rapport d'évaluation. Aussi, dans la perspective de ces rapports, il nous semble essentiel que le texte précise qu'ils devront également faire préalablement l'objet d'un débat au sein de l'assemblée délibérante initiatrice. Ce débat permettra notamment d'informer l'ensemble des membres de l'EPCI de la façon dont a été mise en oeuvre cette expérimentation voire, si besoin, de corriger d'éventuelles difficultés. Quel

l'article 1 en précisant qu'à la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport présentant les communes participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de cette Le présent amendement vise à préciser le champ de cette évaluation intermédiaire de l'expérimentation. Elle doit porter, en particulier, sur les résultats de la formation complémentaire dispensée aux agents de la police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire, l'efficacité de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État

l'intérieur. Les observations des collectivités territoriales et des établissements publics participant à l'expérimentation doivent être annexées à ce rapport.

et exigence, quand il s'agit d'une compétence régalienne. Mais peut-être aurez-vous plus d'enthousiasme pour celui-ci, qui traite de l'atterrissage de l'expérimentation. Le Sénat vient d'adopter une loi sur la simplification de l'expérimentation, disposant qu'à l'issue d'expérimentations de transferts de champs de compétences autorisés par la loi, l'expérimentation peut-être

expérimenter cette compétence. Cela signifie que l'on va imposer à des collectivités qui n'ont pas exprimé cette volonté un transfert de compétence. Il me semble que, dès lors que nous abordons le sujet de l'expérimentation, il faut en étudier l'atterrissage.

qu'aux communes volontaires pour accepter cet élargissement de compétence.

au moment de l'atterrissage. Cela étant, nous savons tous que, dans cinq ans, le législateur aura toute latitude pour définir les modalités du moment. Pour autant, rien n'empêche le législateur d'aujourd'hui

la qualité de la loi, d'écrire aujourd'hui, dans un article de loi, quelque chose qui prétendrait contraindre le législateur dans cinq ans. Madame Gatel, puis-je vous faire observer que le texte sur l'expérimentation auquel vous faisiez référence est un texte de loi organique

la création d'une police municipale relevant de la seule volonté d'un conseil municipal. On ne peut donc imposer à une collectivité ni la création ni le dimensionnement de sa police municipale.

et sur la manière dont on doit apprécier le terme de différenciation. En introduisant, dans ce débat important, l'amendement que, je l'espère, nous allons voter dans un instant, nous émettons un signal d'alarme montrant que nous sommes très vigilants sur ce sujet, nous ne ferons pas des expérimentations dans n'importe quelles conditions et qu'on ne mettra pas en oeuvre le droit à la différenciation dans n'importe quelles conditions.

s'il décide du maintien et de la généralisation des mesures prises à titre expérimental, doit subordonner cette extension des prérogatives judiciaires des agents de police municipale à la demande expresse des communes.

Un exemple de verbalisation AFD : si le Sénat et l'Assemblée nationale valident le fait que les policiers municipaux peuvent mettre des AFD pour consommation de stupéfiants,

municipaux. Aujourd'hui, la police municipale ne peut pas constater le squat de locaux qui n'appartiennent pas à la commune.

qui ne relèvent pas de la police municipale. Il faut évidemment lutter très fortement contre les squats. La police nationale et la gendarmerie doivent être au rendez-vous, à la demande des procureurs de la République le cas échéant. La loi Wargon permettra d'améliorer considérablement la situation, mais les policiers municipaux n'ont pas les moyens d'enquête judiciaire leur

et plus de la moitié d'entre eux- 57 % exactement - sont dotés d'une arme à feu. Alors que le délitement de la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité se poursuit à chaque bavure policière à chaque absence de sanction des infractions commises par ces agents, et alors que l'image de la police se dégrade de manière exponentielle depuis les manifestations des gilets jaunes, nos polices municipales, faisant fi de ces constatations, sont de plus en plus armées. Cela ne va aucunement dans le sens de de la restauration de la confiance nécessaire afin que l'action des forces de sécurité se déroule dans les meilleures conditions possible et que celle-ci soit respectée par tous. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires affirme son opposition au virage sécuritaire caractérisé par une police municipale d'intervention armée et offensive, présente sur la majorité du territoire. Le maintien de l'ordre devrait être considéré comme une prérogative régalienne de l'État, quand la police municipale devrait assurer un rôle de police de proximité, une police du quotidien. Le présent amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires tend ainsi à prévoir un moratoire sur le désarmement de la police municipale et une étude d'impact sur la relation entre police municipale et citoyens. Quel

se dispenser d'écouter ? Les relevés d'infraction qui sont prévus plus tôt à l'article 1 se font sous l'autorité hiérarchique du maire.

Je ne partage pas l'explication de texte que vient de faire M. Richard. « Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire » signifie que le maire continue à avoir une autorité hiérarchique sur le directeur et sur le chef de service de police municipale.